vous est donné de votre mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

La procédure d'examen accélérée ainsi proposée, qui réduit par deux les délais dans lesquels les organisations syndicales majoritaires peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de l'accord, ne permet pas de garantir un délai

article de manière à aboutir à un relèvement réel des minima de branche au niveau du SMIC. Au 17 juin 2022, sur les 171 branches du régime général, 120 affichaient une grille salariale comportant au moins un coefficient inférieur au SMIC en vigueur après sa revalorisation de mai dernier, comme l'a souligné notre collègue Fabien Gay. Par cet amendement, nous proposons de retirer le bénéfice des réductions de cotisations sociales aux branches dont les minima restent en dessous du SMIC durant plus de six mois. Le Gouvernement n'entend pas augmenter significativement le SMIC, d'ailleurs partagée par la majorité sénatoriale. Nous assistons à une précarisation de la société et des salariés, le tout dans un contexte d'inflation très élevée. Il n'est pas possible de vivre correctement avec le SMIC ; alors, imaginez ce qu'il en est en dessous ! Les travailleurs et travailleuses concernés ne cessent de le crier pour être entendus.

des délais de recours fixés aux organisations syndicales et professionnelles. Nous parlons là de quelques jours seulement, mais ce sont des jours utiles pour que ces organisations puissent faire valoir un éventuel droit de recours.

au regard de notre objectif partagé de retour à l'emploi et de valorisation du travail, dans l'intérêt des personnes, de la société en général et de nos finances publiques en particulier. Nous venons d'examiner les articles 1 à 4 . Les mesures de revalorisation du travail resteront assises sur le volontarisme et l'initiative des employeurs et des branches. En revanche, les mesures proposées dans cet article vont s'appliquer de manière globale et indifférenciée. Mon intervention a pour objet

ce qui constitue le plus haut taux d'inflation depuis 1985. Ce taux augmente chaque mois de manière constante : 4,8 % en avril, 5,2 % en mai, 5,8 % en juin ... À ce rythme, l'inflation pourrait atteindre 8,4 % au début de l'année prochaine. Tout cela a de quoi inquiéter nos concitoyens. concitoyens. Face à cette inflation galopante, j'entends le Gouvernement s'enorgueillir de protéger les Français. Or il s'agit surtout, dans cet article 5, d'une prise en compte anticipée de l'inflation sur les pensions et les prestations sociales. monsieur le ministre, que ce que vous donnez aujourd'hui sera déduit des revalorisations à venir auxquelles les Français auraient eu droit : ce n'est pas un cadeau, c'est une avance En raison du niveau de l'inflation, cette revalorisation de 4 % ne redonnera pas réellement du pouvoir d'achat à nos concitoyens et atténuera à peine la perte qu'ils ont subie dans ce domaine. Tel sera notamment Le minimum vieillesse continuera d'être inférieur au seuil de pauvreté- ce n'est pas tolérable ! Plus de 10 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. La crise sanitaire est venue aggraver la situation de millions d'hommes et de femmes. Je pense notamment aux familles monoparentales, qui peinent à boucler leur budget au point de grossir les rangs des structures d'aide alimentaire. Compte tenu de cette situation, la revalorisation anticipée des pensions et des prestations sociales ne peut en aucun cas être acceptée pour solde de tout compte : il nous faut impérativement conserver la possibilité de clauses de revoyure avant janvier 2023, pour un réel soutien à nos concitoyens et une réelle protection de leur pouvoir d'achat.

interrogation porte sur le financement de ces mesures. Monsieur le ministre, l'ensemble de ce projet de loi coûtera 20 milliards d'euros. Les mesures spécifiques de cet article vont coûter 4 milliards d'euros à la sécurité sociale et 2,6 milliards d'euros au budget de l'État.

Pourtant, nous ne sommes pas avares d'idées, et il me semble que certaines pourraient être mises en oeuvre.

-, les revenus liés à l'AAH sont intégrés dans la base des revenus pris en compte pour le calcul de l'éligibilité au RSA, ce qui n'est pas juste, notamment dans les cas de transfert

le retour à l'emploi. D'ailleurs- pardonnez-moi pour cette parenthèse -, je pense que la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité lorsqu'elle a attribué 575 euros par mois à un allocataire du RSA

aux entreprises et aux employeurs pour augmenter la valeur du travail ! Oui ! Ne venez pas nous faire la leçon sur la revalorisation du travail pour baisser le montant des prestations de gens qui survivent à peine avec quelques centaines d'euros par mois, alors que vous refusez la revalorisation du travail

la cohésion nationale. Mais ce n'est pas en abondant cette fausse représentation d'un lien direct entre les revenus de remplacement et le désamour du travail que nous réglerons ensemble le problème. Par ailleurs, la meilleure façon de creuser l'écart entre les revenus de remplacement et les salaires, c'est d'augmenter les salaires.

nous, la revalorisation, c'est par le travail qu'on l'obtient, mes chers collègues. Sinon, c'est de la monnaie de singe

Le texte fondateur de notre République, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle les devoirs ne sont cités qu'une fois : dans le préambule. Les droits

et les prestations sociales. En effet, comme cela a été souligné, si la revalorisation anticipée des retraites et des prestations sociales est plus que nécessaire, elle ne sera pas à la hauteur. Elle demeure en

Surtout, l'Insee anticipe d'ores et déjà une inflation à presque 7 % en septembre. Ce rythme resterait ensuite compris entre 6,5 % et 7 % d'ici à la fin d'année. Par conséquent, conséquent, cet amendement vise à procéder à une réévaluation du coefficient appliqué par le présent article, afin de le corriger éventuellement à la hausse dans le cas où l'inflation progresserait encore fortement.

des bénéficiaires des prestations, allocations et aides individuelles, dont le montant est à réévaluer avec l'inflation. Si l'on peut considérer qu'une partie des mesures gouvernementales, comme la revalorisation anticipée des pensions de retraite et des prestations familiales ou le triplement du plafond de la prime dite Macron, représentent un soutien bienvenu aux ménages, force est de constater qu'elles demeurent ponctuelles et inférieures à l'inflation. En outre, la revalorisation anticipée prévue pour juillet vient seulement réduire la perte de pouvoir d'achat sur la seconde partie de l'année et ne remédie pas au problème de sous-indexation des prestations sociales, qui a déjà réduit le pouvoir d'achat des plus pauvres pendant la première moitié de l'année. Les mesures de revalorisation des prestations sociales prévues dans ce texte, à hauteur de 4 %, doivent être considérées d'ores d'ores et déjà comme une sous-indexation desdites prestations alors que l'inflation prévue par l'Insee atteindra 5,2 % en 2022. Il convient donc de faire toute la lumière sur les pertes de pouvoir d'achat subies par les plus fragiles d'entre nous, ceux qui travaillent dur ou qui ont cotisé toute leur vie pour leur retraite.

Les amendements que je vais présenter visent avant toute chose à réaffirmer les problématiques sociales et économiques de la Corse, lesquelles appellent des réponses structurelles d'autant plus fortes que la crise, si elle nous impacte tous, touche l'une des régions les plus pauvres du territoire, où près de 19 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Si elles ont vocation à être débattues dans le cadre du processus de négociation engagé, ces questions peuvent et doivent être anticipées dans le cadre de nos débats parlementaires afin de répondre à l'urgence de la situation. Ce premier amendement vise à prendre en compte dans les mesures portant sur l'augmentation du pouvoir d'achat prévues dans le les spécificités de la Corse telles qu'elles ont été énoncées lors de la conférence sociale pour le respect des droits fondamentaux des citoyens de Corse dans le domaine économique et social, qui s'est tenue le 23 mai 2022 à Bastia.

Enfin la reconnaissance ! C'est la reconnaissance que l'AAH n'est pas une prestation sociale comme les autres : la reconnaissance du droit d'aimer sans perdre ses droits reconnaissance, enfin, de l'autonomie financière des personnes en situation de handicap même si, nous le savons, pour vivre dignement, cette allocation n'est pas suffisante. Il en aura fallu, du temps

dans cet hémicycle. Puis, à la suite de la pétition la plus importante jamais reçue en ces murs, cette proposition de loi a été remise sur la table. Bravo aux personnes en situation de handicap, bravo aux associations de n'avoir rien lâché Il aura fallu que le Président de la République soit pris à partie devant les caméras pour que l'instant d'émotion filmé prenne force de loi. Alors oui, nous ne boudons pas notre plaisir de voir enfin reconnues les personnes handicapées. Mais que de temps perdu ! Presque cinq ans,

C'est l'affirmation même que retarder la jouissance des droits de nos concitoyens et concitoyennes permet d'économiser les postes de fonctionnaires nécessaires pour accélérer cette mise en oeuvre. Néanmoins, nous voterons l'article 5 . La parole

Certes, cette mesure a un coût, de l'ordre de 400 millions d'euros en année pleine. Mais il s'agit de défendre une grande cause, des valeurs hautement symboliques.

revalorisée de plus de 100 euros, pour monter jusqu'à 904 euros par mois, soit une augmentation de pouvoir d'achat de près de 12 % pour 1,2 million de bénéficiaires. La déconjugalisation de l'AAH constitue donc une véritable mesure de justice sociale, attendue par nos concitoyens en situation

Nous connaissons les difficultés techniques à surmonter et nous savons pouvoir compter sur la mobilisation du Gouvernement et de l'administration pour que cette réforme prenne corps le plus rapidement possible. Cette mesure entraînera un gain de pouvoir d'achat pour 160 000 personnes. Quant au dispositif transitoire prévu par l'article, il permettra de trouver toutes les solutions adéquates pour les quelque 45 000 personnes qui seraient perdantes avec la déconjugalisation simple.

Je souhaiterais, pour ma part, soulever une autre problématique en matière de prestations sociales. Je veux vous interpeller, monsieur le ministre, au sujet des femmes vivant seules avec leurs enfants et bénéficiant de prestations sociales.

à leur indépendance financière et, vous en conviendrez, proprement injustifiée. Elle fait peser sur le nouveau couple une pression inopportune, car le nouveau compagnon, je le rappelle, n'est pas le père des enfants. Il y a là une certaine forme d'injustice que je tenais à mettre en lumière, qui s'apparente à une forme

Je vous invite donc à regarder de près l'idée d'une déconjugalisation de certaines prestations sociales- je pense tout particulièrement à l'allocation de rentrée scolaire. Très

et le sujet de l'autonomie financière des personnes handicapées reste sur la table. Nous attendons une grande loi en matière d'autonomie depuis de nombreuses années. Une promesse a été faite, et nous avons la volonté d'aller plus loin en matière d'autonomie.

Ainsi, un maire qui est aussi paysan retraité ne peut prétendre à la revalorisation que cette loi entraîne. En effet, il continue à cotiser en tant que maire, et cette loi prévoit qu'il faut avoir liquidé l'intégralité de ses droits à la retraite pour bénéficier de la revalorisation. Nous soutiendrons d'autant plus cet article qu'il s'agit d'une des rares mesures de progrès et de justice sociale de ce texte. Au bout du compte, il s'agit d'exprimer notre reconnaissance aux agriculteurs, aux chefs d'exploitation qui s'engagent dans la vie de leur village. vie de leur village. Dans mon département, le Pas-de-Calais, 750 communes sur 890 comptent moins de 2 000 habitants. Ce sont donc 750 maires ruraux qui s'investissent chaque jour. Parmi eux, un grand nombre sont d'anciens agriculteurs. Nous sommes leurs obligés, en tant que représentants des collectivités et de la ruralité. Le groupe CRCE votera donc cet article. Très bien

parole est à Mme Corinne Féret. Face à la plus forte inflation recensée depuis trente-sept ans, accentuée par la guerre en Ukraine et un contexte géopolitique incertain, les Français nous demandent d'être à la hauteur des enjeux. La détresse sociale grandissante que nous constatons chaque jour dans nos territoires nous oblige à agir rapidement et efficacement. Le pouvoir d'achat est une préoccupation légitime de nos concitoyens. La réponse à apporter aux difficultés qu'ils éprouvent doit couvrir les principaux volets de notre économie. Cet amendement vise qu'une conférence nationale du pouvoir de vivre, réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, de l'Insee, ainsi que des acteurs qualifiés du monde associatif, soit créée et mise en place avant la fin de l'année 2022, 2022, pour faire le point sur l'efficacité des mesures issues du présent projet de loi et proposer rapidement de potentiels ajustements. Outre les mesures d'urgence, cette nouvelle structure de dialogue social et de concertation serait chargée d'élaborer des mesures structurelles à mettre en oeuvre pour soutenir le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Français. Ce travail ferait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement. Il faut bien comprendre, mes chers collègues, que la période nous appelle à changer nos façons de penser et d'envisager l'avenir. Nous devons passer du pouvoir d'achat au pouvoir de vivre, car c'est bien de cela dont il s'agit : se loger, se nourrir, se déplacer, se vêtir, vivre dignement de son travail, se former, avoir accès à une vie sociale et culturelle ... La mise en place de cette conférence nationale du pouvoir de vivre est plus que jamais légitime et d'actualité.

Je n'en ferai pas, et je souhaite que, sur toutes les travées de cet hémicycle, nous soyons conscients de l'extrême gravité de la situation énergétique française. Tous les rapports qui émanent de Bruxelles nous annoncent un hiver terrible. Le coût de l'électricité en France pourrait être jusqu'à cinq fois supérieur à ce que l'on observera dans d'autres pays européens. C'est une fragilité incroyable du système français. Cette fragilité vient de notre incapacité à anticiper depuis plusieurs décennies, avec une espèce de nostalgie pompidolienne de la France, de son parc nucléaire,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2019, ici même, dans cet hémicycle, nous avions voté la fermeture des quatre centrales à charbon

! « Le réel, c'est quand on se cogne », disait Lacan. Aujourd'hui, le réel, ce sont nos 29 réacteurs nucléaires en carafe et un mix énergétique complètement déséquilibré qui nous pousse au bord du gouffre.

Afin de protéger juridiquement les dispositifs d'accompagnement social inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mis en oeuvre sur le site de la centrale Émile-Huchet de Saint-Avold,

pourquoi, je le redis, nous devons avoir un débat ici, au Parlement, sur l'avenir de l'opérateur EDF et sur la politique énergétique. M. Patrick Pouyanné, dont ne peut pas dire qu'il soit communiste ou écologiste, appelle lui-même

Mme Raymonde Poncet Monge. La guerre en Ukraine met sérieusement en danger nos approvisionnements en gaz, et ce alors que 5 millions de ménages, il faut le rappeler, sont déjà en situation de précarité énergétique en France.

l'étape de renouvellement des CDD de dix-huit mois. Pour toutes ces raisons, nous proposons par cet amendement de supprimer la possibilité de conclure dès le départ des CDD jusqu'à trente-six mois- on s'inscrit presque directement dans cette perspective

d'autant plus impérieuse que la situation internationale met désormais en péril l'approvisionnement en énergie de la France pour cet hiver.

Le salaire moyen des salariés concernés s'établissait autour de 4 500 euros nets. Ils seront réembauchés de manière temporaire avec une augmentation de 5 % par mois, assortie d'une prime

en exemple pour la particularité de son mix énergétique, qui, par des prises de décision remontant à de nombreuses années, a favorisé les énergies renouvelables.

donc qu'il ne faut pas opposer les modèles de production. Dans le cadre des discussions que nous aurons sur la future programmation pluriannuelle de l'énergie, il faudra adopter

On parle tout le temps de l'Allemagne ; aujourd'hui, les contrats qui s'y négocient pour le pic de consommation de l'hiver sont trois fois moins chers qu'en France. Donc, l'Allemagne, avec

et de confiance aux travailleurs de ce secteur, dont nous allons avoir besoin pour sortir de la crise actuelle, il faut voter l'amendement n° 193 ! Je mets

Merci

et agents publics. Régie par le décret du 24 octobre 1985 et une circulaire du 12 mars 2001, cette indemnité vise à compenser le niveau élevé des loyers dans les zones tendues. Son montant est dérisoire, voire indécent. Par ailleurs, le dispositif actuel devrait être élargi à certaines zones, notamment les zones frontalières, qui en sont pour l'heure exclues. Je pense, en particulier, au Pays de Gex dans l'Ain ou aux zones frontalières de Haute-Savoie. La situation est à ce point tendue dans ces zones qu'elle met en péril la continuité du service public dans l'enseignement, la santé, la police. Aujourd'hui, par exemple, des candidats au concours préfèrent renoncer à son bénéfice plutôt que d'exercer dans ces zones, trop chères.

J'ai par ailleurs appris que le comité interministériel de la transformation publique avait décidé, en février 2021, d'une mission sur l'attractivité territoriale de la fonction publique prenant prenant en compte ces questions indemnitaires et de logement. Je souhaiterais donc savoir où en est cette mission et quelles en sont les conclusions. Ne faudrait-il pas un rapport plus spécifique sur le sujet ? La parole

Nous considérons que la question reste posée. Elle est d'une brûlante actualité ! La crise du logement, même du logement cher, dans notre pays ne pourra se traiter avec des « mesurettes ». Le logement, qui reste le premier poste de dépenses des ménages, plus particulièrement de leurs dépenses préengagées,

Cette hausse bénéficierait essentiellement aux multipropriétaires, qui détiennent les deux tiers du parc de logement des particuliers. Pire, les ménages propriétaires d'au moins cinq logements, s'ils ne représentent que 3,5 % de la population, possèdent 50 % des logements mis en location.

Je vous remercie,

dans cet hémicycle, la question du logement, du pouvoir d'achat et de l'accès au logement à un prix modéré est une priorité du Gouvernement. Je suis saisi

pour favoriser la construction de logements sociaux. On ne peut évoquer la question du pouvoir d'achat dans les outre-mer sans parler du prix des logements.

Face à la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie, il est nécessaire de protéger les plus précaires en établissant des mesures visant à limiter la hausse du prix des loyers pour les locataires. À ce titre, nous appelons le Gouvernement à aller au-delà de la revalorisation à 3,5 % des APL afin de permettre à leurs bénéficiaires de faire face à la hausse des charges locatives résultant de l'augmentation du prix de l'énergie.

lequel est formellement en dehors de la discussion commune qui va suivre, vise à proposer un plafond de 1 % dans le parc locatif privé. Il n'y a pas de raison de distinguer le parc social du parc privé. Une hausse de 3,5 % sur un an conduit, selon toute vraisemblance, à ne répercuter que la moitié de la hausse de l'inflation. Les bailleurs prennent donc toute leur part de l'effort. Le Gouvernement a trouvé un compromis équilibré

La part du loyer dans les charges contraintes est de plus en plus élevée pour les ménages les plus pauvres. Selon la Fondation Abbé Pierre, le loyer représente 36 % des dépenses contraintes des ménages les plus précaires après redistribution. Selon l'Insee, l'ensemble des charges contraintes représentent 41

Encore une fois, l'inflation se répercute davantage sur les plus modestes, qui ont vu leur pouvoir de « solvabilisation » des APL chuter depuis 2017 à la suite de plusieurs contre-réformes, dont la baisse de cinq euros restera la plus scandaleuse.

Le nombre d'amendements que nous avons collectivement déposés sur cet article 6 témoigne de la nécessité de contenir l'évolution des loyers. Pour la plupart des locataires, ce taux d'effort devient difficilement tenable. Sur ce point essentiel de la maîtrise de l'évolution du coût du logement, qui pèse très lourd dans le budget des ménages, il faut rappeler qu'aucune mesure durable n'a été engagée pendant le quinquennat précédent aucune intervention, pas même pour maîtriser l'envolée des prix du foncier ; refus d'une généralisation de l'encadrement des loyers, ne serait-ce dans les zones tendues affaiblissement des acteurs essentiels, notamment ceux du logement social ... Ces choix se sont traduits par une baisse historique de la construction de logements abordables. Le Gouvernement se contente aujourd'hui d'une mesure d'urgence ponctuelle, provisoire et très insuffisante pour protéger le pouvoir d'achat et l'accès au logement des citoyens. Il ne s'agit pas ici d'opposer, comme on peut l'entendre, propriétaires et locataires. L'enjeu est de maintenir de maintenir un équilibre soutenable pour tout le monde. Or il faut bien admettre que la pression du coût du logement pèse aujourd'hui davantage sur les locataires. À cet égard, l'étude d'impact rappelle que les propriétaires ont bénéficié d'une dynamique de prix très positive ces dernières années,

Les prix ont ainsi augmenté de 25 % en cinq ans. De surcroît, les petits propriétaires ne détiennent que 8 % du parc locatif, tandis que 3,5 % des ménages propriétaires d'au moins cinq logements détiennent la moitié du parc locatif privé.

des personnes les plus modestes. Alors que le loyer est le principal poste de dépenses contraintes des ménages, le soi-disant « bouclier logement » proposé par le Gouvernement est largement insuffisant pour protéger le pouvoir d'achat des Français, déjà confrontés à une hausse du prix de l'énergie, des carburants et de l'alimentation. Le Gouvernement nous explique que le plafonnement à 3,5 % est équilibré. Monsieur le ministre, vous avez appelé à une nouvelle méthode pour légiférer, dans un esprit de compromis et de coconstruction. Or les associations et les représentants de locataires n'ont visiblement pas été consultés. On attend des propriétaires qu'ils s'engagent fortement dans la transition énergétique, ce que nous pouvons entendre. Mais ils sont soutenus financièrement par l'État dans cet effort. Les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale pour moduler l'évolution des loyers dans la limite de 1,5 % ou de 2,5 %, selon que les locataires

des propriétaires. Rappelons que les loyers des uns sont les revenus des autres et que de ces revenus dépend notamment la capacité des propriétaires à procéder aux travaux de rénovation énergétique exigés par la loi Climat et résilience et assortis d'interdiction de louer.

d'une réfection d'électricité ou de la création d'un ascenseur. Ces augmentations ne sont pas indues. Ces investissements ne peuvent être réalisés à fonds perdu par les bailleurs. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

Le projet de loi propose une revalorisation des APL de 3,5 %. Or un gel des loyers ou un plafonnement inférieur de l'IRL auraient été plus efficaces pour protéger les locataires, dont le loyer représente le principal poste de dépense. Tout cela n'est pas cohérent. Rafraîchissons notre mémoire pour justifier la baisse de cinq euros des APL au début du quinquennat précédent, le Gouvernement pointait leur effet inflationniste. Ainsi, les quelques euros de cette revalorisation iront directement dans la poche du bailleur sans condition et, plus grave encore, ne suffiront pas à combler la potentielle augmentation de loyer. Une fois encore, la protection des bailleurs, et notamment des fameux 3,5 % des ménages détenteurs de 50 % du patrimoine, se fera au détriment des ménages les plus modestes. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent d'instituer un gel de la hausse des loyers dans les zones tendues, là où le marché de l'immobilier demeure spéculatif.

lorsque le loyer n'a pas été révisé depuis plus d'un an ; lorsque le loyer est manifestement sous-évalué ; et lorsque des travaux importants ont été réalisés. Il est toutefois impossible

nationale, permettant une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers en fonction de critères géographiques. Il s'agit d'introduire une triple dérogation pour mieux prendre en compte les situations spécifiques à chaque territoire.

et la hausse des loyers et des charges est moins élevée que sur le reste du territoire. Un plafonnement de la revalorisation des loyers à 1,5 % y serait donc légitime, d'autant que le revenu fiscal par unité de consommation médian y est faible.

objectifs : coût de la vie plus élevé qu'en France métropolitaine, loyers représentant un poids plus substantiel dans les dépenses totales des ménages en outre-mer et taux de pauvreté plus élevé qu'en métropole. cet amendement tend à introduire une modulation dans le plafonnement de la variation des loyers à hauteur de 1,5 % pour la collectivité de Corse, afin de mieux prendre en compte l'insularité et ses répercussions sur le niveau de vie des habitants.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages, le Gouvernement a souhaité plafonner à 3,5 % la variation de l'indice de référence des loyers jusqu'en juin 2023. À l'Assemblée nationale, les députés ont introduit une modulation

Elle a également estimé que l'inflation et le montant des loyers dans les outre-mer étaient comparables à ce que l'on observait dans l'Hexagone, et que cette mesure ne se justifiait donc pas. Mes chers collègues, je ne vous apprendrai rien : il est toujours délicat de brandir le respect de l'égalité quand on parle des territoires ultramarins, parce qu'il existe des inégalités de traitement, dont on trouve des exemples jusque

Cet amendement tient donc compte de ces inégalités en visant à plafonner à 2,5 % la variation de l'IRL dans les outre-mer et à revenir ainsi au texte adopté à l'Assemblée nationale.

Je vais aborder successivement les cas des ZRR et de la Corse puis des outre-mer, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles la commission a pris la décision de supprimer les exceptions introduites par l'Assemblée nationale. Le point commun à toutes ces dispositions est qu'elles visent à faire varier le plafond de hausse des loyers en fonction de considérations locales, alors que l'indice de référence des loyers utilisé est national et s'applique à tous ces territoires.

l'avis du conseil départemental ou de l'assemblée de Corse et un arrêté préfectoral. En outre, ils reposent pour partie sur des données inexistantes ou parcellaires. Enfin, ils aboutiraient à la définition d'un très grand nombre de plafonds des loyers dans chaque département, voire à un niveau infradépartemental, puisqu'ils ouvrent la possibilité d'une modulation du plafond retenu. Cela pose un problème d'intelligibilité de la loi et d'insécurité juridique au détriment des locataires comme des bailleurs, et cela pose également un vrai problème de constitutionnalité. Il nous faut mettre en balance cette grande complexité avec leur durée de vie, limitée à une année.

les loyers outre-mer représentent plutôt une part moins importante dans les dépenses des ménages qu'en province, et l'inflation y a été plus contenue qu'en métropole.

élue de Saint-Barthélemy, où les loyers atteignent des niveaux vertigineux, et je mesure la charge que peut représenter ce poste budgétaire pour un ménage et les risques sociaux que cela emporte, particulièrement dans cette période de hausse des prix. Cette compétence appartenant à la collectivité, le présent dispositif ne s'y appliquera pas, bien entendu. Le rapport sur le logement social outre-mer, que j'ai eu l'honneur de présenter avec mes collègues Victorin Lurel et Guillaume Gontard, me permet de connaître l'ampleur des besoins et des enjeux de ce secteur. Aussi, je suis convaincue que la proposition de plafonnement que nous examinons contribuera à préserver le pouvoir d'achat et à protéger les locataires, notamment les plus fragiles. Le taux différencié de 2,5 % correspond à un compromis tenant compte des revenus des locataires comme des bailleurs. Nous devrons toutefois demeurer attentifs aux difficultés de financement de l'entretien des bâtiments, que les bailleurs sociaux anticipent et sur lesquels ils ont d'ores et déjà alerté. La cherté de la vie pesant essentiellement sur les denrées alimentaires, peut-être aurait-il fallu cibler davantage ces dépenses. En tout état de cause, nous devons être pragmatiques et limiter l'augmentation à 2,5 %. Cela contribuera à contenir l'accroissement du poids des charges fixes de nombreux ménages, dans les collectivités où 80 % des 80 % des populations sont éligibles à un logement social, pour 15 % de bénéficiaires. Au-delà de l'urgence, en écho aux recommandations du rapport précité, le plafonnement de l'augmentation des loyers rappelle l'urgence de disposer d'évaluations statistiques régulières et précises.